J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire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

Partant de ce principe, nous devons renforcer les dispositions législatives qui nous permettent, au sein de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes, du ministère de l'intérieur et du ministère de la justice, de mieux lutter contre la fraude fiscale et contre toute forme de fraude.

La question médiatique, peut-être même parfois anecdotique, plus que profonde, du « verrou de Bercy » occupera sans doute une partie de nos travaux. Le Gouvernement n'a pas souhaité l'intégrer dans le texte

service, dirigé par un magistrat- en l'occurrence, une magistrate -et qui dépend du ministre de l'action et des comptes publics, même s'il est évidemment autonome, puisqu'il ne peut être saisi que dans le cadre

Je suis prêt à examiner les dispositions que vous évoquez, monsieur le rapporteur- peut-être faudra-t-il les affiner si vous permettez que nous ayons une discussion sur ce point. Vous aurez constaté qu'il n'y a pas d'amendement de suppression concernant, notamment, la TVA

Mais ils sont aussi parfois, et souvent en premier lieu, confrontés à des contrebandiers, des fraudeurs, des malfaisants, on peut le dire, qui les rudoient avec une certaine énergie. Or la loi ne permet malheureusement pas de sanctionner comme il se doit ceux qui ne se plient pas aux contrôles des douaniers.

Enfin, par l'article 10, nous souhaitons mettre en avant le travail très important des douaniers, en aggravant les sanctions contre ceux qui entravent leur action. Deux derniers points sont en débat. L'article 11 évoque la liste des paradis fiscaux, des trous noirs fiscaux, en bref, des pays qui ne jouent pas le jeu que la France souhaite mener, à l'instar de certains autres pays. Aussi, nous devons ici prendre des engagements.

Viendra le moment, dans un an et demi, où les choses seront constatées. C'est ainsi que l'Union européenne a construit sa liste noire. Sans doute les choses sont-elles

dans le passé, nous avons eu un désaccord avec la Commission européenne sur ce point. Mais l'augmentation du prix du tabac, assumée par le Gouvernement et qui porte ses fruits, vise à lutter très fermement contre ce qui pourrait s'apparenter à un laisser-aller en

dans la prise de conscience des enjeux liés à la fraude et l'évasion fiscales, avec une mise en tension des finances publiques. Il en a sans doute résulté une volonté de lutter contre les phénomènes d'évitement de l'impôt ; cela s'est imposé comme un impératif économique et social, qui mobilise bien sûr à la fois les pouvoirs publics

applicables. Il doit s'entendre, selon l'exposé des motifs lui-même, comme le « pendant » du « droit à l'erreur », que le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance tend par ailleurs à reconnaître.

: le cumul entre une sanction administrative et une sanction pénale doit être réservé aux cas les plus graves. Et le Conseil constitutionnel a énuméré un certain nombre d'éléments prouvant la gravité des faits.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux tout d'abord vous remercier de m'avoir confié la tâche de rapporter, au nom de la commission des lois, une partie de ce projet de loi, une première expérience d'autant plus enrichissante qu'elle répond à une attente citoyenne forte. En effet, s'il y a encore quelques années les fraudeurs fiscaux n'étaient considérés que comme faisant défaut aux intérêts financiers d'un État, aujourd'hui ces manoeuvres frauduleuses sont perçues comme portant une atteinte directe à l'effort de probité et de solidarité que tout Français, personne privée ou morale, doit avoir envers ses concitoyens. Il est donc nécessaire que le système actuel évolue. S'il convient de renforcer la sanction d'un contribuable qui se soustrait sciemment à ses obligations contributives, il y a consensus à ne porter devant la justice que les affaires les plus emblématiques et pour lesquelles l'exemplarité de la sanction pénale, avec la publicité qui s'y attache, présente un intérêt majeur. Pour ce faire, ces règles doivent être transparentes et légalisées, et c'est tout le sens du travail qui a été mené au Sénat. La commission des finances a délégué au fond à la commission des lois l'examen des articles 1, 8 et 9, et la commission des lois s'est saisie concomitamment pour avis de l'article 5. Aussi, je vous ferai part des conclusions de l'étude approfondie que la commission des lois a menée sur ces quatre articles. En ce qui concerne l'article 5 relatif à la publicité des condamnations pour fraude fiscale, plus communément appelée le, la commission des lois estime le dispositif proposé est satisfaisant, en ce qu'il permet de rétablir une règle de condamnation dissuasive, qui se concilie avec le principe d'individualisation des peines. Elle entérine également en l'état l'article 8, qui traite de l'alourdissement des amendes prévues en cas de fraude fiscale, en les portant au double du produit tiré de l'infraction. La commission des lois juge pertinent l'article 9, qui vise à étendre à la fraude fiscale la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, plus communément appelée le « plaider-coupable sur l'initiative du procureur, permet d'éviter un long procès, sans effacer pour autant la culpabilité de l'auteur, puisque la peine est homologuée par le président du tribunal de grande instance en audience publique. La commission des lois veut même aller plus loin, puisqu'elle propose d'introduire deux outils complémentaires à la disposition des juges. Nous proposons, en premier lieu, d'inscrire la jurisprudence dans la loi. Depuis 2008, la Cour de cassation considère que le parquet peut engager des poursuites sur le fondement du blanchiment de fraude fiscale, le blanchiment étant considéré comme un délit distinct de la fraude. L'objet de notre amendement est donc de sécuriser les procédures engagées depuis une dizaine d'années sur la base de cette jurisprudence. En second lieu, dans le même esprit et en lien avec une proposition pertinente de nos collègues députés, Émilie Cariou et Éric Diard, formulée dans leur rapport d'information sur le verrou de Bercy, nous vous proposons d'étendre à la fraude fiscale la possibilité de conclure une convention judiciaire d'intérêt public, la CJIP. CJIP. La conclusion d'une telle convention par une personne morale est possible sur la seule proposition du procureur. Elle implique de verser au Trésor public une amende d'intérêt public et de mettre en oeuvre un programme de mise en conformité. La convention est obligatoirement homologuée par un juge, qui doit également en faire publicité un communiqué de presse. Déjà autorisée pour le blanchiment de fraude fiscale, la CJIP a été utilisée avec succès par le parquet national financier pour traiter certains dossiers. Il est donc cohérent de l'autoriser aussi pour la fraude fiscale. Enfin, la commission des lois a procédé à la suppression de l'article 1, qui vise la création, au sein du ministère du budget, d'un nouveau service à compétence nationale chargé de mener des enquêtes judiciaires en matière de fraude fiscale. Sur ce point, monsieur le ministre, nous avons une divergence forte : si le Sénat a montré sa volonté de « déverrouiller Bercy » dans ses travaux menés au cours des dernières semaines- sa position est d'ailleurs constante depuis des années -, ce n'est certainement pas pour entrer dans une logique de création d'une police de Bercy Depuis 2010, procureurs et juges d'instruction peuvent s'appuyer sur une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, la BNRDF. Dépendant du ministère de l'intérieur, et coadministrée par Bercy, cette brigade associe des officiers de police judiciaire et des officiers fiscaux judiciaires. Elle peut ainsi mettre en oeuvre les techniques d'investigation de la police judiciaire et bénéficier d'une expertise pointue en matière fiscale. Cette brigade, originale par sa mixité de fonctions, comprend environ quarante personnes, qui peuvent s'appuyer sur l'ensemble du maillage territorial de la police judiciaire, soit environ 5 700 personnes. Le Conseil d'État précise dans son avis qu'un second service d'enquête judiciaire fiscale hors du ministère de l'intérieur serait concurrent du premier. Il dit même ne pas comprendre pourquoi, dans un souci de bonne administration, n'est pas retenue l'option consistant à renforcer le service existant. La commission des lois et la commission des finances sont également peu convaincues du bien-fondé de la création d'une nouvelle police, alors que la BNRDF a déjà pour mission de mener des enquêtes fiscales, et uniquement cela. Il nous semble plus sain

Merci

du présent projet de loi, et des amendements qui s'y rattachent, jusqu'après l'article 13. En effet, l'article 9 modifie l'article L. 228 du livre des procédures fiscales. Or plusieurs amendements déposés à l'article 13 tendent à proposer une nouvelle rédaction de ce même article, voire à l'abroger. Aussi convient-il d'examiner l'article 13

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Didier Rambaud.

un texte qui s'inscrit dans la continuité du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance et dans un ensemble de mesures qui donnent un sens à l'action du Gouvernement. de la responsabilité et de l'émancipation, pour permettre à chacun d'avoir une chance de lutter contre les rentes et de punir ceux qui trichent. Le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui n'intervient pas en réponse à une affaire ou à un scandale, comme cela a pu se produire sous les majorités précédentes, mais comme une réponse pragmatique à un combat qui prend encore plus de sens dans un pays qui arrête de surréglementer, qui cesse d'imposer à ses entreprises et à ses citoyens des obstacles qui n'existent pas à l'étranger. Mais ce permis de faire ne signifie pas laisser-faire ! C'est tout l'enjeu du projet de loi que vous présentez, monsieur le ministre. Mes chers collègues, nous avons ici un texte qui apporte une réponse pragmatique à un ensemble de comportements de fraude, ainsi que de nouvelles dispositions qui aideront les services de l'administration à lutter contre ces comportements. C'est le cas de l'article 2, qui renforce les moyens des agents des douanes pour logiciels conçus pour permettre ou organiser la fraude. Les agents auront accès au code source et à la documentation des logiciels en cause. Il s'agit d'une mesure de bon sens, qui répond à un besoin identifié des agents des douanes. le travail de ces derniers est reconnu à travers ce projet de loi, un travail difficile mais ô combien majeur ! Le texte rend plus effectif le droit de communication dont les agents des douanes bénéficient pour la recherche de la fraude douanière et l'établissement de l'assiette des impositions douanières. Certes, comme pour les avancées de l'article 3 sur l'échange et l'ouverture de fichiers à différents métiers, notamment aux assistants spécialisés mis à disposition des juridictions, personne ne félicitera le Gouvernement pour ces mesures, mais elles seront aussi efficaces qu'elles sont attendues par ceux qui travaillent au quotidien contre ce qui mine notre pacte républicain. Gardienne d'un temps long au seul bénéfice de l'intérêt général et de la Nation, notre assemblée doit se réjouir de mesures qui ne sont prises ni dans l'émotion ni dans la réaction. Ce texte est un texte pragmatique, pragmatique, mais pas seulement. En réalité, la philosophie sur laquelle il repose a deux jambes : pris comme un tout, les mesures proposées allient pragmatisme et exemplarité. 6, l'introduction du en droit français ou encore l'automaticité de la peine complémentaire de publication en cas de fraude fiscale. Voilà deux mesures nécessaires et complémentaires à la confiance qui est accordée aux entreprises et aux particuliers. Ceux qui travaillent en respectant les règles ne peuvent supporter l'impunité face aux comportements déloyaux. Enfin, ce texte prévoit de nouvelles voies juridictionnelles utiles, comme l'extension de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à la fraude fiscale, qui permettra une réponse pénale plus rapide et plus efficace. Le plaider-coupable en matière de fraude fiscale, c'est un gain de temps dans le traitement des procédures de fraude fiscale, une réparation plus rapide pour les parties civiles et une répression plus effective, mieux acceptée et exécutoire de plein droit. Mes chers collègues, face à ce texte, nous devons faire le choix de l'efficacité. Tout d'abord, j'appelle le Sénat à la raison pour qu'il réintroduise l'article 1, supprimé par la commission des lois. Au regard de l'importance du sujet pour nos concitoyens, comment peut-on s'opposer à la création d'un nouveau service de lutte contre la fraude ? Comment peut-on croire que les postes qui allaient être créés seront créés ailleurs ?

Acceptons de créer un nouveau service et évaluons plus tard son action et son efficacité. Ne nous privons pas de moyens supplémentaires pour lutter contre la fraude ! Par ailleurs, ne cédons pas au corporatisme facile : je pense au souhait de certains de supprimer l'article 7, qui, non seulement nuirait à la logique d'ensemble du texte, mais supprimerait également une mesure jugée efficace et dissuasive par les experts du droit. En outre, mes chers collègues, j'entends souvent un Sénat critique à l'égard des textes longs et complexes. Or nous avons là un texte initial court, articles, dont l'architecture est claire. Respectons ce paquet de mesures. Le Parlement aura le temps de les évaluer plus tard, de les améliorer et de les compléter au besoin.

Le groupe La République En Marche suivra donc l'évolution du texte à travers les discussions que nous aurons ensemble. Notre groupe soutiendra les mesures qui complètent le texte, comme ont pu le faire nos collègues rapporteurs de la commission des lois et de la commission des finances, et s'opposera aux mesures d'affichage, inapplicables ou qui réduiraient de fait l'efficacité de la réponse face à la fraude, que cette réponse soit administrative ou pénale. Notre groupe souhaite également rappeler l'excellent travail de nos collègues députés membres de la mission d'information commune sur les procédures de poursuite des infractions fiscales. C'est parce que nous respectons le droit d'amendement de nos collègues parlementaires de l'Assemblée nationale que nous ne soutiendrons pas les mesures qui se réfèrent aux conclusions de cette mission, conclusions qui ne contiennent aucune proposition légistique, je tiens à le rappeler. Il en va de même pour l'article 13, qui nous donnera néanmoins l'occasion d'une discussion dans l'hémicycle, plus propice au débat démocratique que dans la presse ! La parole

Monsieur le ministre, lorsque le Gouvernement auquel vous appartenez a annoncé en début d'année son plan de lutte contre la fraude, certains se sont pris à rêver du grand soir fiscal. Enfin ! Voilà un gouvernement proactif qui s'attaque au dossier de l'évasion fiscale, sans y être poussé par un nouveau scandale révélé par la presse ou les lanceurs d'alerte. C'est dire si nous attendions avec une certaine impatience vos propositions. À la lecture de votre projet de loi, nous voulons vous dire d'emblée que nous restons sur notre faim Ce texte est encore fortement marqué par une forme d'indulgence à l'endroit des fraudeurs fiscaux. Il reste très modeste dans ses ambitions, se contentant pour l'essentiel d'aménagements à la marge, de modifications cosmétiques et d'un renforcement des sanctions fiscales administratives. Il s'inscrit avant tout dans une volonté globale de marginaliser la poursuite pénale des auteurs de délits fiscaux, la légitimité d'un traitement principalement administratif de la fraude fiscale et de tenter de rendre politiquement acceptable le maintien du « verrou de Bercy », qui constitue pourtant une spécificité difficilement défendable et tout à fait inacceptable pour l'ensemble de nos concitoyens. Dans ce texte, il n'y a pas un mot sur les grands groupes du numérique, pas un mot sur une liste crédible des paradis fiscaux en Europe et dans le monde, pas un mot non plus sur les lanceurs d'alerte, qui ont pourtant joué un rôle essentiel ces dernières années dans les révélations de scandales d'évasion fiscale, très peu de mots, enfin, sur la dimension internationale du sujet. Aux premières annonces du début d'année, à grand renfort de tambours et trompettes médiatiques, vous avez annoncé la création d'une police fiscale, une nouvelle équipe de trente agents, cinquante à terme. C'était la mesure phare de ce projet.

Quoi que l'on puisse dire, ces suppressions d'emplois ont des conséquences directes sur les conditions d'exercice du contrôle fiscal. Regardons un peu les chiffres de Bercy pour l'exercice 2017 : une baisse de 2 % des vérifications de comptabilité pour l'année, baisse de 5 % des droits et pénalités des opérations répressives. Tandis que le nombre d'entreprises a augmenté de 15 % entre 2010 et 2016, le nombre de vérifications n'a cessé de diminuer. Pendant que l'on parle de lutte contre la fraude fiscale, le taux de couverture des services du contrôle fiscal sur les entreprises a reculé de 22 % en quelques années

techniques et financiers à tous les services existants, afin qu'ils puissent encore augmenter leur efficacité. Monsieur le ministre, l'article 11 de ce projet de loi prévoit d'intégrer la liste des paradis fiscaux de l'Union européenne à la liste française. Cette disposition pourrait prêter à sourire si elle ne traitait pas d'un sujet aussi grave pour les finances publiques. Pour mémoire, rappelons la maigreur de la liste française, qui comporte sept États : le Botswana, Brunei, le Guatemala, les Îles Marshall, Nauru, Niue et le Panama, ce dernier État ayant été rétabli en catastrophe dans la liste en avril 2016, au lendemain des révélations fracassantes des « Panama papers », par le consortium international des journalistes d'investigation.

Pourtant, la planète « évasion fiscale » y tourne très bien. Depuis 2016, année de la révélation de l'affaire dite « LuxLeaks », qui dénonçait ces accords fiscaux très avantageux pour les grands groupes, le Grand-Duché de Luxembourg a conclu 599 accords fiscaux de ce type,

d'une exception française qui, au fond, institue une justice à deux vitesses. On nous rétorque invariablement que le dispositif actuel est plus efficace en termes de montants et de rapidité. Cela reste bien évidemment à vérifier. Quand une présomption se fait jour, elle ne peut être établie qu'en recourant à des moyens coercitifs qui, dans un État de droit, ne peuvent être autorisés que dans le cadre d'une procédure judiciaire. C'est ainsi qu'il peut arriver que des indices ne soient ni traités ni transmis à la justice. Pour véritablement rétablir la confiance chez nos concitoyens, l'heure est à la transparence et à la justice. Mes chers collègues, M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, déclarait à l'Assemblée nationale le 6 novembre dernier, au lendemain des nouvelles révélations des « Paradise papers » que « l'évasion fiscale est une attaque contre la démocratie Il est très regrettable que ces propos n'aient pas été suivis d'effets véritables. Depuis trente ans, des politiques de fiscal ont été menées par certains pays, y compris au sein de l'Union européenne. Ces politiques trouvent leur origine dans la liberté complète de circulation des capitaux, décrétée dans les années quatre-vingt, et érigée en véritable dogme depuis. Une guerre sans merci s'est alors développée pour attirer les capitaux. Dès qu'un État assouplit sa législation fiscale, les capitaux bondissent vers le pays d'accueil. Je ne suis pas de ceux qui se résignent à cette injustice ! Dès lors qu'il y a un impôt, certains cherchent à s'en affranchir. C'est tout à fait inacceptable ! La différence entre évasion et fraude fiscales me laisse toujours un peu pantois. lors que vous élaborez des systèmes particulièrement opaques pour ne pas payer l'impôt, qu'un certain nombre de manoeuvres sont accomplies, qu'une ingénierie est mise en place dans une très grande opacité, les jurisprudences et la perception que l'on en a aujourd'hui pourront évoluer ... un jour. Mes chers collègues, les élus, la République, sont au pied du mur pour réaffirmer ici le primat de l'intérêt général. Ce texte en l'état ne nous y conduit pas. Puisse le débat en enrichir la portée ! La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, madame la rapporteur, mes chers collègues, dans son esprit, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui peut être directement relié au projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public. Le droit à l'erreur que ce dernier texte prévoit d'introduire au bénéfice du contribuable de bonne foi rend plus que nécessaire, en contrepartie, le durcissement de la répression de la fraude fiscale, dont l'ampleur offense la République et l'honnêteté de chaque citoyen. Si nécessaire et cohérent fût-il, le projet de loi initial examiné par la commission des finances du Sénat n'était pas parfait, et encore moins complet. C'est pourquoi je tiens à saluer le travail de la commission des finances et de son rapporteur, grâce à qui la copie du Gouvernement a été substantiellement nourrie et améliorée. Le texte comporte désormais une vingtaine d'articles, là où la version initiale n'en comptait que onze. Je ne prendrai qu'un exemple : les apports de la commission des finances concernant le renforcement de la lutte contre la fraude sur internet, avec l'instauration inédite d'un régime de responsabilité solidaire des plateformes en ligne pour le paiement de la TVA due par les vendeurs qui y exercent leur activité. Le montant de cette fraude est estimé en France, pour les seules ventes de biens matériels, à plus de 1 milliard d'euros. Il faut développer les contrôles. Nous espérons que le régime, qui a été introduit voilà deux ans outre-Manche et qui a déjà fait ses preuves, prospérera à l'issue du texte, avec votre avis bienveillant, monsieur le ministre. Il me semble toutefois que ce projet de loi peut aller plus loin et, avec lui, la lutte contre la fraude fiscale. C'est pourquoi je soumettrai à votre appréciation deux amendements visant à aider l'administration à renforcer son accès à l'information auprès des experts-comptables et de leurs collaborateurs, qui sont si souvent les premiers témoins de la fraude fiscale. Je profite également du temps qu'il m'est donné pour saluer la commission des lois et le travail de son rapporteur, Nathalie Delattre, qui a permis d'enrichir le texte. Je pense notamment à l'introduction de l'article 9, qui permet d'entériner la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt et, donc, d'écarter l'application du « verrou de Bercy » en cas de poursuites pour blanchiment de fraude fiscale. Nous aurons à reparler du « verrou de Bercy » dans les heures qui vont suivre. C'est pourquoi je ne m'attarderai pas davantage sur le sujet. Je terminerai en soulignant les apports au texte de ma collègue Nathalie Goulet, apports que nous soutiendrons. Mes chers collègues, ce projet de loi revêt à nos yeux une importance particulière, qui tient à la sensibilité politique, médiatique et sociétale du sujet. En effet, lorsque la fraude n'est pas correctement appréhendée et réprimée, l'édifice fiscal et social est compromis. Il nous revient collectivement de préserver et d'encourager l'honnêteté, c'est-à-dire garantir de punir. Le texte, sous réserve des modifications qui seront apportées lors de son examen à venir, agit en ce sens.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, nous nous retrouvons pour débattre du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, contre les fraudes.

dans cette lutte. Plein de bonnes intentions, ce texte ne peut cependant être qualifié de « grand texte » : avant son examen en commission, il n'apportait aucune avancée significative en ce qui concerne la fiscalité des plateformes d'économie collaborative, par exemple.

Nous saluons avec satisfaction le fait que la commission des finances, dans une belle unanimité, ait amélioré les dispositions fiscales applicables aux plateformes collaboratives et proposé dispositif clair pour lutter contre la fraude à la TVA sur internet. Nous espérons que le Sénat, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, sera entendu au cours de la navette parlementaire qui suivra. S'agissant des paradis fiscaux, nous regrettons que la liste de ces derniers soit aussi peu élargie à des pays dont les pratiques fiscales s'apparentent à un véritable. Le texte de la commission va dans le bon sens, mais ne va pas encore assez loin. Il est temps que la France reprenne la main, puisque la Commission européenne a fait montre de son impuissance. Enfin, concernant le verrou de Bercy, nous sommes surpris de voir le rapporteur continuer à communiquer sur sa suppression. En effet,

Le texte de la commission prévoit certes un aménagement, mais largement insuffisant. Il s'agit d'automatiser la transmission de certains dossiers au parquet. Parfait ! Ces dossiers devront correspondre à des critères. Très bien ! En effet, personne ne souhaite envoyer 15 000 dossiers devant des tribunaux, car ils seraient alors engorgés. Mais ces critères sont très restreints, trop restreints et, surtout,

son dossier automatiquement transmis. Il n'est pas raisonnable que les critères définis soient cumulatifs. De très nombreux dossiers vont encore passer entre les mailles du filet, dans la droite ligne du manque de transparence qui caractérise la situation actuelle. Nous regrettons vivement que, pour une partie de nos collègues, la lutte contre la fraude se limite à l'encaissement des droits et pénalités pour les malchanceux qui se sont fait prendre. Nous regrettons aussi que la poursuite pénale n'apparaisse, dans ce cadre, que comme un moyen de pression pour amener le contrevenant à négocier. La convention juridique d'intérêt public est par ailleurs l'aboutissement de cette logique qui tend à faire de la justice une simple gestionnaire et à vider la procédure pénale de sa substance. C'est la raison pour laquelle nous n'y sommes pas favorables.

Parallèlement, une mission d'information relative à la fraude fiscale a été créée à l'Assemblée nationale et a été citée. Le rapport de cette mission et ses propositions ont recueilli l'approbation de tous les partis politiques y ayant participé. Tous ont reconnu l'excellence du rapport. La mission a défini le chemin à suivre et nous devons, devant cette unanimité, répondre présent et ne pas proposer de fausses solutions qui ne seraient que de la communication politique. Les conclusions de la mission Cariou répondent parfaitement aux enjeux, qui ne se limitent d'ailleurs pas à la suppression du verrou de Bercy. Vous retrouverez, dans nos amendements, des propositions de traduction dans la loi de ses recommandations. La levée du verrou de Bercy doit permettre la transmission aux parquets de tous les dossiers correspondant aux fraudes fiscales aggravées. Nous proposerons de définir dans la loi les critères non cumulatifs qui détermineront l'envoi automatique Nous avons constaté que plusieurs sénateurs de différents groupes politiques présentent des amendements identiques. Nous espérons que cette démarche permettra de faire vivre au Sénat les propositions issues de la commission de l'Assemblée nationale. « verrou de Bercy » est une condition indispensable pour un dispositif antifraude efficace et transparent, mais elle n'est pas suffisante.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, madame le rapporteur pour avis, mes chers collègues, « la fraude est à l'impôt ce que l'ombre est à l'homme OEuvres complètes ! C'est ce que disait Georges Pompidou ! La fraude serait une sorte de fatalité, un mal que nous serions impuissants à éradiquer.

S'y ajoutent la fraude aux cotisations sociales, que la Cour des comptes estime à 20 milliards d'euros, et la fraude à la TVA, qui représente au moins 14 milliards d'euros par an en France, d'après la Commission européenne. Pourtant l'impôt est ce qui fonde la citoyenneté, le vivre ensemble, la participation de chacun à la vie de la Nation. Les articles XIII et XIV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen rappellent cette exigence une contribution commune est indispensable » et « tous les citoyens ont le droit [ ...] de la consentir librement ». La fraude sape ces fondements républicains de notre société et affaiblit le consentement à l'impôt. Face à la fraude, on peut être fataliste, répéter que « la fraude est à l'impôt ce que l'ombre est à l'homme », ou alors, on peut agir. On peut renforcer notre arsenal préventif et répressif pour l'adapter aux évolutions de la société. C'est ce que fait la France depuis plusieurs années

Ce projet de loi, sans être révolutionnaire, pose une pierre supplémentaire à cet édifice de longue haleine. Il apporte des « petites révoltes », comme vous l'avez dit précédemment, des aménagements bienvenus à nos dispositifs de lutte contre la fraude. Tout abord, ce texte renforce les pouvoirs de contrôle et de sanction des douanes, tout en favorisant les échanges d'information entre les administrations. Ensuite, et c'est peut-être sa plus grande originalité, il prévoit de nouvelles sanctions à l'égard des fraudeurs et il réforme notre arsenal répressif. L'article 6 du projet de loi permet à l'administration fiscale, sous certaines conditions, de rendre publiques les sanctions administratives qu'elle prononce à l'encontre des personnes morales, au titre de certains manquements particulièrement graves. Cette introduction du anglo-saxon dans notre tradition juridique doit s'accompagner de garanties fortes, à la mesure du risque « réputationnel » encouru. Notre commission des finances y a pourvu en prévoyant que seules les sanctions définitives pourront faire l'objet d'une publication. En outre, la liste française des États et territoires non coopératifs s'enrichit des juridictions figurant sur la liste du Conseil de l'Union européenne. Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, les critiques dont fait l'objet ce type de listes, notamment celle de l'Union européenne. On pourrait la muscler encore par l'insertion des juridictions à haut risque identifiées par le Groupe d'action financière, le GAFI. Ce sont des États qui facilitent le blanchiment de la fraude fiscale internationale et le financement du terrorisme. Ils méritent, à ce titre, une vigilance approfondie. Je ne m'attarderai pas sur les ajouts de notre commission des finances relatifs à la lutte contre la fraude à la TVA sur les plateformes en ligne. Ce sont des recommandations que le Sénat formule depuis longtemps et qui permettraient de nous inspirer des meilleurs exemples étrangers pour récupérer plus de 1 milliard d'euros par an. En revanche, notre commission a saisi l'opportunité que vous lui aviez offerte à propos du « verrou de Bercy » : elle propose un dispositif équilibré avec trois critères cumulatifs qui entraînent le dépôt obligatoire par l'administration d'une plainte pour fraude fiscale. Nous aurons certainement des débats très nourris- je l'ai compris -sur cette question et sur la place respective du parquet et de l'administration.

Le régime actuel fait coexister deux procédures parallèles dont la cohérence n'est pas assurée. Nous en avons eu la preuve il y a quelques jours encore avec l'annulation de la mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale d'un milliardaire russe, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre.

du prisme de l'idéalisation du parquet, car quoi qu'il arrive l'opportunité des poursuites, contrairement à ce que certains semblent croire, existera toujours, qu'elle soit le fait d'un spécialiste au sein de

Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte tel que complété par notre commission des finances est un texte équilibré, qui permet des avancées législatives certaines. Nous devrons donner les moyens à la direction générale des finances publiques, la DGFiP, et aux douanes de le mettre en pratique, en utilisant plus largement des techniques nouvelles, comme le « » ou l'intelligence artificielle. Dans la compétition entre les fraudeurs et le régulateur, où les fraudeurs essaient d'avoir en permanence une longueur d'avance, il est de notre responsabilité de veiller à ce que les armes de l'État soient toujours les plus affûtées, les plus rapides et les plus précises possible.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, madame la rapporteur, mes chers collègues, le présent projet de loi s'inscrit dans la lignée des projets adoptés sous les quinquennats précédents et visant à répondre à la problématique de la fraude fiscale, mise en lumière, trop souvent, par une série de scandales, et dont le préjudice pour les recettes fiscales de l'État par le Sénat en 2012 à un montant compris entre 30 milliards et 50 milliards d'euros par an. J'ai entendu, monsieur le ministre, que vous organiseriez une grand-messe à la rentrée pour objectiver le chiffre : espérons qu'il fasse référence nous invitez ... Vous l'êtes ! Il s'agit donc d'un enjeu de finances publiques, mais il s'agit également d'un enjeu sociétal : le consentement à l'impôt peut être raisonnablement remis en cause par l'explosion des scandales de fraude fiscale, encore faut-il qu'il y ait consentement à l'impôt.

Ce projet de loi apparaît par ailleurs comme la contrepartie du projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public, actuellement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, dont la mesure principale est l'instauration d'un droit à l'erreur pour les contribuables. Indulgence pour l'honnête contribuable, sévérité pour le fraudeur : c'est un bon équilibre. La partie répressive se traduit dans le projet de loi que nous examinons aujourd'hui par une série de mesures, utiles pour certaines, sans être pour autant révolutionnaires. Il s'agissait, en premier lieu, de créer une nouvelle police fiscale dépendante de Bercy. Notre commission des lois a jugé cependant cette mesure largement inopportune. largement inopportune. Nous estimons en effet qu'il eût été plus judicieux de renforcer les moyens de l'actuelle BNRDF, ... Oui ! ... comme l'a très bien expliqué Nathalie Delattre. Exactement ! Évitons, monsieur le ministre, une nouvelle guerre des polices, créons plutôt un deuxième bureau, car il a fait ses preuves en son temps. Il s'agit, en second lieu, d'introduire une procédure de « plaider-coupable » pour les infractions de fraude fiscale, mais aussi de publier les noms des plus gros fraudeurs et de sanctionner les intermédiaires financiers coupables de montages financiers frauduleux ou « abusifs », terme que nous jugeons d'ailleurs trop flou. Ce projet de loi sera aussi l'occasion pour le Gouvernement de réformer le « verrou de Bercy » grâce au Sénat, maintenant que l'Assemblée nationale a compris l'ensemble de Vous avez souhaité avancer sur le « verrou de Bercy » lors de l'examen du texte qui nous occupe aujourd'hui, je vous en remercie. Notre commission des finances a fait des propositions sur ce point, j'y reviendrai dans quelques instants. Je souhaiterais tout d'abord rappeler que le Sénat suit de près les questions de fraude fiscale depuis plusieurs années déjà. En juillet 2012, un rapport de notre collègue Éric Bocquet fut publié dans le cadre d'une commission d'enquête sénatoriale présidée par Philippe Dominati. En octobre 2013, un second rapport d'Éric Bocquet, ... Tout aussi excellent ! ... ... ... fut publié à l'initiative d'une commission d'enquête sénatoriale sur le rôle des banques, présidée par François Pillet. Il faut

Actuellement, un groupe de suivi de la commission sur la fraude et l'évasion fiscales travaille également sur le sujet de la fraude. Le Sénat a adopté à plusieurs reprises, souvent à l'unanimité, des mesures contenues dans le rapport de 2017, mais notre assemblée, hélas ! n'a pas été suivie par l'Assemblée nationale. Comme le rapporteur Albéric de Montgolfier, dont je tiens à saluer la constance sur ces sujets, je me félicite du fait que la vertu pédagogique de la répétition ait fait évoluer le Gouvernement, d'une part, et, nous l'espérons, l'Assemblée nationale, d'autre part. Il s'agit de l'obligation pour les plateformes d'économie collaborative de transmettre au fisc les revenus de leurs utilisateurs. Jusqu'à présent, les plateformes n'avaient l'obligation de ne communiquer le montant annuel des revenus qu'à leurs seuls bénéficiaires et de rappeler à ces derniers les règles fiscales et sociales applicables afin de les inciter à les déclarer. Si la commission des finances a depuis longtemps prôné des mesures encourageant la fiscalisation des revenus sur les plateformes en ligne, elle a cependant toujours estimé qu'un abattement était nécessaire. Une franchise de quelques milliers d'euros par an semble préférable à une fiscalisation au premier euro, afin d'exonérer les petits compléments de revenus occasionnels permettant de « boucler des fins de mois », à distinguer d'activités dégageant des recettes plus substantielles et professionnalisées, relevant de la fraude. C'est pourquoi notre groupe soutient l'adoption d'un abattement forfaitaire de 3 000 euros, qui avait déjà été adopté à l'unanimité par le Sénat dans le projet de loi de finances pour 2018, avant d'être rejeté, encore une fois, par l'Assemblée nationale. De la même façon, nous soutenons l'interdiction, pour les plateformes en ligne, d'effectuer des versements à leurs utilisateurs sur des cartes prépayées. Ce système de cartes permet en effet de rendre « invisibles » aux yeux du fisc les revenus perçus par les utilisateurs. Notre commission s'est également intéressée depuis plusieurs années au cas spécifique de la fraude à la TVA. Nous vous demandons, de ce fait, monsieur le ministre, que les dispositions que nous avons adoptées à l'unanimité en commission soient conservées dans le texte final.

entre des vendeurs particuliers, professionnels ou non, et des acheteurs en ligne. Or les vendeurs professionnels situés dans des pays étrangers ne transmettent souvent pas de numéro de TVA à ces plateformes et en conséquence ne paient pas de TVA, ce qui leur permet d'afficher des prix inférieurs

Pour remédier à cette situation, la commission des finances, sur l'initiative de notre rapporteur général, a souhaité que le numéro soit obligatoirement collecté par les plateformes. À défaut, ces dernières doivent être solidaires fiscalement si des vendeurs coupables de fraude à la TVA sont détectés par l'administration et qu'il s'avère qu'aucune mesure n'a été prise par la plateforme. Ce dispositif est inspiré du système britannique qui a fait ses preuves et qui a permis d'augmenter les recettes de TVA L'article 4 adopté par la commission des finances reprend également une mesure envisagée par le Royaume-Uni et déjà adoptée au Sénat à plusieurs reprises. Enfin, notre commission a prévu une solidarité fiscale des filiales françaises des plateformes pour les amendes en cas de non-respect du devoir d'information des utilisateurs quant à leurs obligations fiscales et sociales et en cas de non-transmission au fisc des revenus des utilisateurs, ainsi qu'une solidarité fiscale des filiales françaises des entreprises auxquelles est appliquée l'amende pour manquement au droit de communication non nominatif. La première mesure a pour objet d'éviter que les grandes plateformes, qui sont pour la plupart situées à l'étranger, ne s'affranchissent des obligations prévues à l'article 4, alors même qu'elles disposent de plusieurs filiales en France. La seconde mesure vise, de la même façon, à obliger les filiales françaises des plateformes en ligne à transmettre des informations non nominatives à l'administration fiscale en les rendant solidairement responsables du paiement des amendes. Cette obligation d'information incombe, en effet, aux sites en ligne depuis 2015, mais elle est peu appliquée quand ceux-ci ont leur siège dans un pays tiers. Venons-en maintenant au sujet légendaire du « verrou de Bercy Notre commission des finances a fait des propositions qui, assurément, permettent d'atteindre un équilibre entre la nécessité de l'efficacité et la nécessité de la transparence, reprenant les pistes que j'avais tracées voilà deux mois à cette tribune. En effet, lorsqu'il y a quelques semaines j'ai rapporté la proposition de loi de notre collègue socialiste Marie-Pierre de la Gontrie renforçant l'efficacité des poursuites contre les auteurs d'infractions financières et supprimant le « verrou de Bercy », j'avais mis en garde contre les conséquences d'un transfert brutal de tous les dossiers de fraude fiscale à l'autorité judiciaire. Les risques d'engorgement des tribunaux, de perte d'expertise et de perte de confidentialité sont réels. Le temps de l'impôt est le temps de l'économie, qui n'est pas le temps de la justice. Il y a là un risque majeur. Toutefois, j'avais insisté également sur la nécessité d'encadrer davantage le système afin de le rendre parfaitement transparent et contrôlable. J'avais invité les fonctionnaires de Bercy à ne pas avoir peur de la transparence eu égard à leur probité. Ainsi j'avais prôné, avant le rapport Cariou, que les critères de sélection des dossiers par Bercy et la commission des infractions fiscales, aujourd'hui définis par une circulaire, soient redéfinis par la loi. Tel est l'objet du nouvel article 13, introduit dans ce projet de loi par notre commission des finances. Ce système de critères transparents, car définis par la loi, entraînerait donc obligatoirement le dépôt par l'administration fiscale d'une plainte pour fraude fiscale auprès du parquet. Ces critères sont cumulatifs

l'administration devra aller devant le parquet, qui, comme l'a souligné à juste titre mon collègue Capus, pourra toujours demander à se saisir d'un dossier, même si les deux critères cumulatifs ne sont pas remplis. Ainsi, le parquet reste maître des poursuites. Cette réforme du « verrou de Bercy » n'est peut-être pas la suppression que vous attendiez, le verrou étant trop souvent fantasmé. En tout état de cause, nous garantissons l'efficacité en matière de recouvrement, ce qui est le plus important. Les dossiers les plus substantiels seront confiés à l'autorité judiciaire et les dossiers les moins importants pourront faire l'objet d'un traitement plus rapide, la répartition des dossiers étant fondée sur des critères clairs et contrôlés par la représentation nationale. Pour conclure, le groupe Les Républicains votera ce projet de loi tel qu'il a été amélioré et enrichi par les travaux de notre Haute Assemblée.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, madame la rapporteur pour avis, chère Nathalie, mes chers collègues, ce projet de loi relatif à la lutte contre la fraude a été déposé devant notre assemblée le 28 mars dernier. Après le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance examiné en début d'année en première lecture, et que nous allons bientôt réexaminer en nouvelle lecture, ce texte se présente comme son pendant répressif, comme cela est clairement expliqué dans l'exposé des motifs : « Si, face à la complexité de notre système de prélèvements fiscaux et sociaux, il peut arriver au contribuable de bonne foi de commettre erreur ou oubli, appelant de l'administration un traitement bienveillant, le fait de se soustraire sciemment à ses obligations contributives doit être poursuivi avec la plus grande efficacité, et sévèrement sanctionné ». La fraude fiscale coûterait entre 60 et 80 milliards d'euros par an à l'État, soit environ 20 des recettes fiscales brutes. Ce n'est pas rien ! La fraude la plus importante concerne la TVA. Viennent ensuite l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu.

Il faudrait ajouter entre 40 et 60 milliards d'euros par an du fait de l'optimisation fiscale agressive, je serais même tenté de dire très agressive. Ces chiffres sont obtenus par extrapolation à partir des cas de fraude identifiés par l'administration fiscale, que cette fraude soit intentionnelle ou non. Ils ne correspondent pas au montant effectivement redressé. Enfin, la fraude sociale au sens strict- fraude aux prestations et minima sociaux -ou au sens large- fraude au droit du travail, à l'assurance maladie du fait du salarié ou de l'employeur -existe,

En matière de détection, le projet vise à faciliter l'échange de données entre administrations concourant à la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières, et la transmission d'informations par les plateformes d'économie collaborative. En matière d'appréhension de la fraude, elles renforcent les moyens d'investigation. Enfin, en matière de sanction, les dispositions complètent et alourdissent l'arsenal existant, notamment dans une logique plus large de publicité- c'est important -, mais aussi par des méthodes inspirées du monde anglo-saxon, comme le. Je reviendrai Je reviendrai plus précisément sur l'article 1 du projet de loi. La commission des lois, par la voix de sa rapporteur, a décidé de le supprimer, estimant qu'il conduisait à créer un doublon avec les services d'officiers fiscaux judiciaires déjà présents au sein du ministère de l'intérieur. En cela, la commission a suivi l'avis du Conseil d'État qui s'était montré plutôt défavorable à cette mesure. mesure. L'article 2 vise à renforcer les moyens dont disposent les agents des douanes pour lutter contre les logiciels dits « permissifs », conçus pour permettre la fraude et la dissimuler, à l'instar de ceux dont bénéficient déjà les agents de la direction générale des finances publiques. L'article 3 renforce l'accès à l'information utile à l'accomplissement des missions de contrôle et de recouvrement des agents chargés de la lutte contre la fraude, notamment en ouvrant aux assistants spécialisés de l'autorité judiciaire l'accès aux fichiers de la direction générale des finances publiques. L'article 4, qui a fait l'objet d'amendements nombreux en commission des finances, précise les obligations fiscales et sociales imposées aux plateformes d'économie collaborative. Le titre II du projet de loi prévoit un renforcement des sanctions contre la fraude fiscale, sociale et douanière, ce qui en fait le volet le plus répressif de ce texte. L'article 5 prévoit prévoit par défaut l'application de la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions de condamnation pour fraude fiscale, aujourd'hui prononcée de manière facultative par le juge répressif. L'article 6 prévoit la création d'une sanction administrative complémentaire des sanctions financières existantes, consistant à rendre publics les rappels d'impôts et les sanctions administratives pécuniaires dont ils ont été assortis, une fois devenus définitifs. L'article 7 crée une sanction administrative de 10 000 euros ou, si le montant est supérieur, de 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable, exclusive des sanctions pénales, applicable aux personnes qui concourent, par leurs prestations de services, à l'élaboration de montages frauduleux ou abusifs. L'article 8 aggrave la répression pénale des délits de fraude fiscale en prévoyant que le montant des amendes puisse être porté au double du produit tiré de l'infraction. L'article 9 vise à ouvrir la faculté au procureur de la République de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le fameux « plaider-coupable », en matière de fraude fiscale. L'article 10 renforce les sanctions douanières applicables en cas d'injures, de maltraitance ou encore de troubles à l'exercice des fonctions des agents des douanes, ainsi qu'en cas de refus de communication des documents demandés. Enfin, l'article 11 complète la liste française des États et territoires non coopératifs en matière fiscale afin qu'elle intègre celle qui a été adoptée par l'Union européenne en décembre 2017. Le texte a été enrichi lors de l'examen en commission de plusieurs dispositions, en particulier l'autorisation la convention judiciaire d'intérêt public- ou encore transaction pénale - en matière de fraude fiscale, à l'article 9. À l'article 11 concernant la liste des paradis fiscaux, les membres de la commission des finances avec sagesse la prise en compte de l'échange d'informations et la mention de critère de la liste européenne des paradis fiscaux. Surtout, le nouvel article 13, au sein d'un nouveau titre nommé « réforme de la de la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale », tend à desserrer le « verrou de Bercy » puisque des dossiers qui rempliront certains critères cumulatifs devront automatiquement être transmis au parquet, qui pourra alors engager des poursuites pénales. Ces différents sujets, qui sont présents dans le débat public depuis des affaires ayant émaillé le précédent quinquennat, ont déjà été abordés lors de l'examen de la loi de 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et de la loi Sapin II. Ils résonnent aussi avec l'actualité et les mesures prises à l'échelle internationale, notamment sous l'égide de l'OCDE, avec l'accord multilatéral de 2016 sur l'échange de déclarations pays par pays et, dernièrement, la convention multilatérale de lutte contre l'érosion des bases d'imposition

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, un débat sur la fraude fiscale de plus n'est jamais un débat sur la fraude fiscale de trop Nous sortons, on l'a déjà dit, du cycle « un scandale, une annonce, un texte ». Néanmoins, ce n'est pas le grand soir de la lutte contre la fraude fiscale, comme vous l'avez vous-même reconnu à la tribune, monsieur le ministre. J'ai déposé avec mon groupe une batterie d'amendements,

en particulier, concernant la liste des paradis et des territoires non coopératifs, comme je l'ai déjà dit à cette tribune et puisque c'est la saison, je vous annonce que je déposerai un amendement sur la réforme constitutionnelle de façon que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales soit inscrite à l'article 34 et qu'enfin le Parlement puisse être associé à l'élaboration de cette liste des territoires non coopératifs,

et le renforcement des sanctions fiscales, administratives, ce texte apparaît comme un renforcement d'un traitement administratif de la fraude fiscale, au détriment des poursuites pénales. L'alibi de l'encombrement présumé des tribunaux ne constitue pas un motif sérieux pour justifier un texte modeste dont le contenu ne correspond pas aux attentes d'une société de confiance. C'est un signal. L'impression qui se dégage, parodiant Cyrano, est que vous vous servez une réforme fiscale

comme rapporteur spécial de la mission « Gestion des finances publiques », j'ai eu à évoquer à plusieurs reprises les objectifs de la direction générale des finances publiques : asseoir, recouvrer, contrôler les impôts. Le projet de loi que vous nous soumettez, monsieur le ministre, entre dans ce dernier objectif : contrôler, contrepartie du consentement à l'impôt et d'un système déclaratif. Il fait suite à de nombreuses dispositions fiscales entrées dans notre droit positif sous le précédent gouvernement. Depuis, les révélations de multiples affaires ont jeté un regard insupportable sur l'évasion fiscale agressive et la fraude fiscale organisée. La réprobation des opinions publiques est à la hauteur des montants éludés. Des dispositions du projet de loi, ainsi que les améliorations apportées par la commission des finances, notamment sur la taxation des plateformes de commerce en ligne, sont de nature à favoriser la lutte contre la fraude. Même si elles mériteraient d'être évaluées par la suite, elles ne peuvent qu'être approuvées par le groupe socialiste et républicain. Elles viennent rééquilibrer les mesures déjà adoptées concernant la redéfinition du contrôle fiscal par l'examen à distance des comptabilités, la limitation de durée des interventions sur place et les mesures d'allégement des contrôles par la reconnaissance du « droit à l'erreur Ce projet de loi n'exonère cependant pas d'une redéfinition des missions de l'administration fiscale encouragée par la Cour des comptes dans son dernier rapport thématique, qui évoque une transformation en profondeur des structures et aborde seulement une administration de services et non l'administration de respect des obligations. Dans un précédent rapport, j'ai évoqué les limites d'une administration de services qui demande beaucoup de moyens humains et matériels alors que la dématérialisation se poursuit. Monsieur le ministre, quelle place dès lors réserver au contrôle fiscal, qui concerne environ 10 000 agents sur les 105 000 que compte la direction générale des finances publiques ? Dans le passé, c'est-à-dire dans l'ancien monde, était revendiquée la sanctuarisation des effectifs du contrôle fiscal. Nous constatons qu'il n'en a rien été puisque 3 000 agents entre 2010 et 2017 ont été supprimés dans ce secteur alors que le nombre d'entreprises soumises à la TVA augmentait ; il est passé de 4 millions en 2008 à 5,5 millions en 2016. L'organisation territoriale en brigades n'a que peu évolué et n'a pas suivi la restructuration des secteurs économiques sur nos territoires. Ainsi, une entreprise a plus de risques d'être contrôlée dans certains secteurs industriels en déclin que dans d'autres qui sont en expansion du fait de la métropolisation de nos territoires. La numérisation et l'informatique, qui conduisent à examiner du bureau les comptabilités, pourraient permettre de transférer le contrôle de secteurs en expansion tout en maintenant une présence territoriale, gage d'un bon aménagement du territoire que le Sénat ne peut qu'encourager. Vous le constatez, au-delà du simple problème des moyens humains, la sélection des dossiers souhaitée par l'administration- 20 % par algorithmes -nécessite la présence, aux côtés d'inspecteurs et de contrôleurs très bien formés, d'informaticiens pour déceler les faiblesses d'une organisation d'un contrôle par trop traditionnel. En ce qui concerne les grandes entreprises, en dépit d'une redéfinition incertaine de l'établissement stable, l'échange de données entre administrations fiscales, douanières, sociales et au niveau international ne peut qu'être positif. Un mot sur la « police fiscale ». Le fonctionnement de la police judiciaire douanière sous le contrôle d'un magistrat est une bonne chose. Nous ne pouvons que regretter la position de la majorité sénatoriale de la commission des lois, qui veut supprimer cette possibilité. Nous avons pu apprécier la complémentarité entre la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, la BNRDF, et la police douanière. Dès lors, un complément d'agents, certes modeste, ne peut qu'être le bienvenu. Leur nombre initial limité devrait évoluer et il conviendrait d'éviter de les prélever sur les effectifs du contrôle fiscal. Vous le comprendrez, la position brillamment exprimée par Sophie Taillé-Polian concernant, notamment, « le verrou de Bercy » doit être complétée par une redéfinition des missions du contrôle fiscal que nous appelons de nos voeux. Car nous sommes conscients de l'ingéniosité fiscale et des moyens toujours renouvelés pour éluder l'impôt, et nous ne souhaitons pas que les mesures proposées ne soient que des effets de communication limités par la suppression annoncée de l', et par le plaider-coupable qui permet d'éviter la sanction judiciaire sous couvert d'efficacité et de rapidité. Monsieur le ministre, vous trouverez notre groupe toujours vigilant sur cette question et favorable à des mesures qui permettent de sanctionner tout autant les « cols blancs » que la petite fraude des particuliers. La parole

pour présenter l'amendement n° 6. L'état actuel de traitement du contentieux fiscal, et notamment la nécessité de sortir du cadre de la loi de 1977, ainsi que l'activité de la commission des infractions fiscales, nous impose de définir de nouvelles règles, plus équilibrées, en matière de procédure contentieuse. Rappelons tout de même que le juge de l'impôt statue selon la technique dite « de l'économie des moyens » : si le contribuable, dans sa contestation, soulève à la fois des moyens de fond et des moyens de forme, et que l'un des moyens de forme permet au juge d'annuler le redressement fiscal, ce dernier rendra sa décision sur ce seul moyen de forme sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. Cela pose le problème de la prise en compte des éléments de fond dans le traitement de l'affaire, chacun en conviendra.

entre contentieux fiscal et traitement juridique de la question, ou le recours prévisible à la reconnaissance préalable de culpabilité qui, par principe, ne risque d'intéresser que les justiciables potentiels ayant quelques moyens de transiger est un peu notre démarche dans cet amendement, dont la rédaction pourrait sans doute être améliorée- on en conviendra -, mais qui présente au moins l'avantage de se positionner sur la voie d'une sécurisation grandissante des procédures, et donc de l'évitement des processus formels et formalistes qui ne règlent pas grand-chose aux dossiers. inhérent à la poursuite de la fraude fiscale est suffisamment complexe pour être respecté. Il n'y a sans doute rien de pire, à notre avis, pour un service fiscal ayant instruit un dossier contentieux avec tout le souci requis, et notamment le souci de l'intérêt général, que de voir ce travail et ses conclusions mis en question au travers d'une transaction discrète aux conséquences assumées., assumées., il importe aussi que le bon droit du contribuable poursuivi puisse être respecté. C'est en ce sens que nous vous proposons cet amendement. Dans le cadre de la réforme des amendes fiscales prévue dans le projet de loi, qui deviennent proportionnelles, fixer précisément le montant des impositions fraudées devient indispensable afin d'assurer l'effectivité de la sanction. C'est le travail du juge de l'impôt, et non celui du juge pénal. Organiser la saisine préjudicielle du juge de l'impôt est donc une priorité à laquelle tend à répondre le présent amendement. La parole

afin d'éviter des cas préjudiciables de divergences de jurisprudence entre le juge de l'impôt et le juge pénal, il est absolument indispensable de prévoir une articulation. Pour l'instant, ce sujet n'est absolument pas traité. On peut constater, lors d'enquêtes pénales pour fraude fiscale, que la procédure est extrêmement déséquilibrée, le ministère public et la juridiction ayant tendance à intégrer la position de l'administration fiscale comme celle d'un expert indépendant, alors qu'il s'agit d'une partie poursuivante. Les principes fondamentaux de l'équilibre de la procédure ne sont donc pas respectés. Afin de rétablir cet équilibre,

pratique, bien souvent, le juge administratif -par le contribuable poursuivi pour fraude fiscale, afin qu'il puisse faire juger rapidement si les impositions contestées sont réellement dues. Cela évitera des divergences et des difficultés d'appréciation entre les deux juridictions

Le juge pénal n'est pas juge de l'impôt, ce qui peut poser des difficultés réelles, notamment par rapport à une sanction qui pourrait être fixée en fonction du montant des droits. Il y a, certes, une possibilité de question préjudicielle, prévue à l'article 386 du code de procédure pénale. La difficulté, c'est que

À chaque audition, monsieur le ministre, j'ai posé la même question et chaque fois on m'a répondu la même chose, à savoir qu'il y avait un problème. Par exemple, un classement sans suite de l'enquête pénale pour fraude fiscale n'a aucune autorité de la chose jugée vis-à-vis du juge administratif, juge de l'impôt, alors même que le procureur de la République, saisi par exemple à la suite d'un avis favorable de la CIF, a déterminé qu'il n'y avait pas de délit de fraude. Ne pensez-vous pas, dans ces conditions, que la loi devrait évoluer pour donner une autorité à l'extinction des poursuites pénales, afin que le juge de l'impôt ne rende pas de décision contradictoire, comme vient de le dire notre collègue, en édictant des pénalités pour mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses ?

c'est justement parce qu'il y a ces critères qu'on évite ces contradictions ! Si on envoyait tous les dossiers, il y aurait évidemment contradiction ... Madame la sénatrice, vous allez surtout permettre à tous les avocats bien intentionnés du monde de gagner du temps. Que fait un avocat ? Il essaie de gagner du temps sur la forme et sur le fond.

mais aussi- avouons-le ! -pour ne pas encombrer les tribunaux avec des dossiers qui ne seraient pas sérieux. Quand on transmet des dossiers, c'est qu'on pense qu'ils sont sérieux, sinon on ne les transmettrait pas ! La DGFiP elle-même considérait sans doute qu'un dossier qui ne va pas jusqu'au bout est un échec.

en contradiction avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Cela concerne peu de cas, mais cette situation est tout de même très choquante : en effet, on apprend en première année de droit que, parmi les éléments constitutifs d'une infraction, il y a certes l'élément intentionnel, mais également l'élément matériel. L'élément matériel,

un combat de toute la société : c'est, bien sûr, l'affaire d'une administration, du politique, de l'exécutif et du législatif, mais aussi, plus largement, celle des citoyens, parce que tout le monde paye l'impôt, qui contribue au fonctionnement de la société dans laquelle nous vivons tous. Mais nous avons nous-mêmes nos principes constitutionnels, selon lesquels, notamment, chacun doit être en mesure de participer à la charge commune à raison de ses facultés, c'est-à-dire de la réalité des revenus qu'il tire de son travail comme de ses biens et de ses avoirs. tend donc à ramener le débat au niveau de l'entreprise, là où tout commence en quelque sorte, pour l'essentiel, qu'il s'agisse de la production de biens et de services, de celle des salaires, revenus essentiels de la population, de l'assiette de la TVA, de l'impôt sur les sociétés, ou encore des cotisations sociales. Nous proposons donc de compléter utilement la base de données en y faisant figurer, au-delà des mouvements financiers, pour les organisations des salariés au sein de l'entreprise, la réalité des relations fiscales entre l'entreprise et l'administration fiscale, sous forme de l'indication des impôts et taxes normalement acquittés et de ce qui resterait de dettes fiscales éventuelles. le sait, l'existence des acomptes de l'impôt sur les sociétés acquittés au fil de l'année budgétaire motive l'absence de telles dettes et engendre plutôt des créances sur le Trésor. Cela posé, les élus du comité seraient par ailleurs délivrés de leur obligation de secret professionnel si l'analyse de ces données permettait, au fil du temps, de déceler ici ou là l'existence d'une fraude fiscale présumée. La commission souhaite le retrait de ces amendements, car elle considère que le droit existant y satisfait. Dans les listes des informations que peuvent obtenir les représentants syndicaux, on trouve les informations sur les investissements, les rémunérations, les flux financiers

la possibilité pour les représentants du personnel de bénéficier d'une protection personnelle, dès lors qu'ils dénoncent des faits constitutifs d'un délit tel qu'une fraude fiscale. Votre amendement, monsieur le sénateur, est satisfait par la loi, sauf à démontrer l'inverse.

Dans le même esprit que le précédent, cet amendement vise à renforcer les droits d'alerte accordés, dans les entreprises, aux instances représentatives du personnel. La plus grande part des dossiers de fraude fiscale concerne des entreprises, et les impôts les plus fraudés sont la TVA et l'impôt sur les sociétés, tandis que la fraude sociale concerne bien plus souvent des cotisations non acquittées que des systèmes de fausses déclarations ou de fraude aux allocations par des particuliers Il est donc évident que c'est à partir de l'entreprise que nous pouvons trouver les voies et moyens d'une lutte préventive efficace contre la fraude fiscale et sociale. Quel est l'avis de la commission ? En abaissant

de fraude fiscale. Tout le monde est d'accord ici pour que la société civile dans son ensemble agisse afin de faire reculer ces manquements réitérés au pacte républicain que peuvent constituer des actes de fraude sociale et fiscale. Nous avons bien conscience, avec cet amendement, que nous partons de l'existant législatif, mais nous souhaitons le renforcer. Dans plusieurs domaines, le législateur a fini par reconnaître quelques vertus à l'action de groupe et a autorisé les associations agréées à ester en justice, avec l'ensemble des droits accordés à la partie civile. L'article 2-23 du code de procédure pénale, largement complété, comme l'ensemble des articles figurant dans cette partie du code, par la loi pour l'égalité réelle et la loi de modernisation de la justice du XXI siècle, prévoit que toute toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes : les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées

les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées à d'autres articles encore dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées ; enfin, les infractions réprimées aussi à plusieurs articles du code électoral. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. Très simplement, on peut donc ester en justice pour combattre le trafic d'influence, le manquement au devoir de probité, le recel ou l'achat de votes lors de consultations électorales. On peut aussi se porter partie civile pour des faits de recel et et de blanchiment, mais pas pour ce qui concerne la fraude fiscale, alors même qu'il s'agit de l'une des préoccupations essentielles des associations non gouvernementales de lutte contre la corruption. Nous vous demandons, au bénéfice de ces observations, mes chers collègues, d'adopter cet amendement qui, nous le reconnaissons une nouvelle fois,

assez différents : dans l'immense majorité des cas, la fraude fiscale n'implique pas la corruption d'un agent public. Or, lorsque la loi permet à une association de se porter partie civile, elle le prévoit toujours pour des infractions en lien direct avec l'objet de l'association. Je le répète, l'objet anticorruption n'est pas celui de la fraude. Ensuite, cet amendement permettrait à des associations de saisir la justice et d'obtenir éventuellement l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits de fraude fiscale,

Le ministère du budget aurait la responsabilité de cette police fiscale, qui pourrait être saisie par des magistrats pour enquêter notamment sur les cas très précis de fraude fiscale,

Je signale que le ministère de l'intérieur, depuis la création de cette brigade, a tout de même changé quelque peu de priorité. Depuis quelques années, notre pays est tout de même très largement concerné par les questions de sécurité et de terrorisme.

Nous avons un service d'enquêtes douanières qui, parce qu'il a l'habitude du fonctionnement de Bercy, pourrait utilement aider cette police fiscale : l'idée n'est pas de les confondre, mais de les mettre l'un à côté de l'autre, en lien. Ce travail montre son efficacité puisque, comme je l'ai évoqué, rien que l'année dernière, le service des enquêtes douanières a effectué à peu près 900 millions d'euros de saisies. de saisies. Il ne s'agit pas d'une guerre des polices ou de supprimer un service pour un autre, il s'agit de compléter l'arsenal que les magistrats auraient sous leur responsabilité, avec des

Je crois qu'il ne faut pas se tromper effectivement sur les missions de cette brigade : elle intervient sur un champ d'enquête bien plus large que les seuls dossiers de présomption caractérisée de fraude fiscale, c'est-à-dire des dossiers où la fraude fiscale n'est qu'un élément de l'affaire. Ce que propose le Gouvernement, et qui vient d'être très bien expliqué par M. le ministre, c'est bien de créer un nouveau service spécialisé dans la fraude fiscale, face au nombre croissant de dossiers complexes. Voilà une proposition plus qu'utile ! Par ailleurs, mes chers collègues, soyons-en conscients : refuser la création de cette police fiscale ne se traduira pas par davantage de personnel au sein de la BNRDF. Quel

tout comme le Conseil d'État, qui a donné un avis défavorable. Il existe déjà au ministère de l'intérieur, on l'a dit, la BNRDF, qui est dirigée par un commissaire de police issu de ce ministère et qui est codirigée par un inspecteur des finances publiques issu de Bercy. La BNRDF est compétente pour enquêter, à la demande du parquet ou d'un juge d'instruction, sur les affaires complexes qui nécessitent des investigations. Le nouveau service que le Gouvernement propose de créer aurait le même champ de compétences que la BNRDF et serait donc un service non pas complémentaire, mais concurrent.

qu'il y six directions à compétence nationale sur le sujet : la direction des vérifications nationales et internationales, la direction nationale d'enquêtes fiscales, la direction nationale de vérification de situations fiscales, la direction des impôts des non-résidents, la direction des grandes entreprises et la direction nationale d'interventions domaniales.

manière assez cohérente, qu'on doit être au sein du ministère de l'intérieur et que Bercy ne doit pas bénéficier de moyens supplémentaires en ce qui concerne les enquêtes.

en présence. Le recours au rescrit permettrait en effet de gérer au mieux les procédures précontentieuses, dans le droit fil de la disposition de contrôle préjudiciel que nous avons évoquée précédemment. C'est d'ailleurs de cette manière qu'une société de presse en ligne, bien connue

divergences. La procédure de rescrit fiscal est là pour éclairer les contribuables en leur permettant de soumettre leur interprétation à l'administration. Si un contribuable n'est pas d'accord avec l'administration, il ne peut pas, en l'état de la jurisprudence du Conseil d'État, contester l'interprétation du fisc devant le juge de l'impôt, car il doit attendre un éventuel contentieux sur le fond. Cela revient à insécuriser les contribuables qui peuvent, le cas échéant, relever de la procédure de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit, voire de poursuites pénales pour fraude fiscale, alors même qu'ils n'ont pas pu encore faire valoir leurs arguments devant le juge de l'impôt.

qui permette d'améliorer significativement les relations entre l'administration et les usagers. La rédaction est précisée par l'établissement d'une suspension de la prescription prescription afin de garantir les possibilités de recouvrement par le Trésor public et d'éviter que des contribuables de mauvaise foi n'abusent de ce nouveau dispositif.

contre un rescrit. Aller plus loin en permettant concrètement de continuer à appliquer sa propre interprétation nous paraît dangereux et pourrait être à l'origine de manoeuvres dilatoires. C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de ces amendements.

La Cour de cassation a en effet saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité le 19 juin 2018. Il s'agissait de faire éventuellement censurer la sanction du délit douanier de blanchiment prévue à l'article 415 du code des douanes. En effet, ce texte, comme il était d'usage précédemment, vise à établir une sorte d'échelle des peines, en lieu et place d'une fixation précise de la peine encourue à raison de l'incrimination. Depuis de nombreuses années, cette manière de légiférer en droit répressif a été abandonnée pour mettre notre droit en conformité avec le principe de nécessité des peines et de liberté du juge à fixer celles-ci. Afin d'éviter une censure potentiellement préjudiciable à la lutte contre la criminalité organisée et la finance criminelle, notamment à vocation terroriste ou à des fins d'évasion fiscale, nous proposons de mettre le code des douanes en conformité avec les principes actuels en supprimant les seuls mots

L'addition totale devrait atteindre 300 millions d'euros à terme. Engie et le Luxembourg contestent. La sanction était attendue depuis l'ouverture d'une enquête à la fin de 2016 contre les pratiques fiscales d'Engie au Luxembourg. Elle a fini par tomber mercredi, en plein rendez-vous- ironie de l'histoire -entre le Premier ministre français Édouard Philippe et le président luxembourgeois de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence,

Les contrôles réalisés par les caisses de sécurité sociale permettent de connecter uniquement les bases des ressources, mais pas celles qui contiennent le patrimoine des personnes qu'elles souhaitent contrôler. La quasi-totalité des prestations servies par les caisses d'allocation familiales le sont sous conditions de ressources. L'article L. 553-5 du code de la sécurité sociale prévoit une évaluation des éléments du patrimoine lorsqu'une disproportion manifeste existe entre le train de vie des allocataires et le montant des ressources qu'ils déclarent. Or les agents de contrôle ne disposent pas des outils nécessaires pour procéder à cette évaluation. L'accès aux bases de la DGFiP rendrait ainsi opérationnel ce qui est prévu déjà par la loi. Pour toutes ces raisons, je vous invite à adopter cet amendement.

impose une grande discrétion, voire une réserve sur ces sujets. Cet amendement vise à permettre à l'administration fiscale de recueillir en direct les informations auprès des experts-comptables et de leurs collaborateurs dans le but d'accroître l'efficience des contrôles. Chaque mois au moins, lors des déclarations de TVA par exemple, les comptables savent très bien qui triche et qui ne triche pas. Ils le savent parce que ces opérations se répètent ou parce qu'elles sont très anormales. Cela ne signifie pas néanmoins que les comptables sont complices. Il faut donc permettre d'exploiter la source de connaissances de la profession en la libérant du secret professionnel dans ce seul cas précis.

? Ces deux amendements portent sur la levée du secret fiscal pour les experts-comptables. Je ne nie pas que les experts-comptables puissent avoir accès à des informations, notamment à des faits constitutifs de fraude fiscale.

a essentiellement une mission de présentation de comptes annuels. Il est lié contractuellement à son client, par un contrat qui peut être résilié à tout moment. Quand un expert-comptable a des doutes sur l'honnêteté fiscale de son client ou qu'il constate des infractions en matière fiscale, il doit se retirer immédiatement de sa mission

en toile de fond, les incidences fiscales que cela peut avoir. Dans 30 % des cas, les bilans des PME sont rectifiés préventivement par le commissaire aux comptes, bien souvent en raison d'infractions fiscales qui sont rectifiées directement. Par ailleurs, si une fraude fiscale est mise en évidence lors de la mission du commissaire aux comptes, il le révélera au procureur de la République et, bien évidemment,

de l'expert-comptable, qui permettent à l'administration fiscale de prendre connaissance d'un certain nombre de choses. Ainsi, l'article L. 86 du livre des procédures fiscales octroie à l'administration fiscale un droit de communication à l'encontre de l'expert-comptable visant ses clients, lui permettant d'obtenir un grand nombre d'informations sur les activités de ses clients. De même, le I

ou des opérations proviennent d'une fraude fiscale. Dans ce cas, l'expert-comptable livre spontanément aux autorités les informations dont il a connaissance. Ces différentes dispositions, qui permettent de lever le secret professionnel, prévoient déjà que l'infraction en cause soit dénoncée le plus rapidement possible.

qui se trouvent dans une situation où il y a un respect du secret professionnel. Les procédures pour lever le secret professionnel sont déjà définies. Pourquoi, du jour au lendemain,

dans la comptabilité du client qu'il doit superviser, il démissionne immédiatement et lui fait une lettre, il dégage sa responsabilité. Pour les inspecteurs des impôts qui sont habitués à voir les bilans régulièrement présentés par tel expert-comptable, quand ils voient que, à tel exercice, d'un seul coup l'expert-comptable s'est retiré, automatiquement ça déclenche une suspicion et ça peut déclencher une vérification fiscale. C'est la première remarque. Ensuite, un amendement tel que celui que présente notre collègue est extrêmement dangereux pour la profession d'expert-comptable. Supposons qu'un expert-comptable dénonce » une présumée fraude fiscale auprès de l'administration ou auprès de la justice et que,, cette fraude ne soit pas avérée, le client concerné pourra alors mettre en cause la responsabilité civile du professionnel pour une révélation non fondée. En revanche, un commissaire aux comptes, qui a l'obligation de révéler toute

les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger au cours de l'année au titre de laquelle doit être déposée la déclaration. Loin de nous l'idée de penser que ces associations ont pour vocation ou habitude de se conformer à des tâches d'optimisation fiscale au-delà de leur objet social ou de leur mission d'intérêt général ou d'utilité publique. Ces informations confirment en général ce qu'il convient de penser de ces associations. En revanche, un doute subsiste sur l'application de ces dispositions aux comptes détenus, mais non mouvementés sur l'initiative du contribuable sur une année donnée, c'est-à-dire ceux sur lesquels il n'a effectué, lui-même, aucune opération de crédit ni de débit durant l'année. L'administration ne pourrait, dans ces cas-là, sanctionner le défaut de déclaration ni mettre en oeuvre la procédure de contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance vie détenus à l'étranger, alors même qu'elle a connaissance d'une telle détention. Afin de clarifier la portée de l'obligation déclarative afférente aux comptes à l'étranger, il est donc proposé de viser l'ensemble des comptes détenus à l'étranger par le contribuable, qu'ils aient été mouvementés ou non durant la période de référence. Dans la plupart des cas, n'en doutons pas, il ne s'agira que d'une simple vérification. Quel est l'avis de la

ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.

Le pacte républicain dont nous évoquons régulièrement les contours et la nécessité passe aussi par les droits et les devoirs de chacun à l'endroit de la sécurité sociale, c'est-à-dire contribuer à son financement par le biais de cotisations en vue de disposer des prestations dues à raison des risques couverts.

La fraude se fait en quelque sorte sur tous les maillons de la chaîne, ce qui donne, soit dit en passant, tout son sens à l'existence d'un réseau des URSSAF suffisamment dense et performant dans ses missions de recouvrement contentieux et à l'existence d'un outil fiscal de proximité digne de ce nom, au plus près du terrain. Pour la commodité du débat, personne ne nous en voudra de procéder à la présentation commune des trois amendements que nous avons déposés à cet endroit du texte. L'amendement n° 75 rectifié vise à augmenter le pourcentage des majorations dues pour les entreprises soumises à un redressement pour retard de paiement réitéré et plus encore pour celles qui ont développé certaines formes de travail illégal. il est important de se souvenir que la lutte contre la fraude sociale n'est pas aussi efficace qu'elle pourrait l'être, si tant est que les URSSAF, d'une part, et que les services de l'inspection du travail, d'autre part, disposaient de moyens plus importants. À moins que la société de concurrence libre et non faussée, ou libre et faussée, selon le point de vue de chacun, n'ait besoin d'un tiers-secteur ne respectant ni règles sociales ni règles fiscales pour continuer d'exister. Les amendements n 77 rectifié et 76 rectifié, quant à eux, tendent à procéder à l'émergence d'un nouveau type de pénalisation de la fraude sociale sous des modalités éventuellement transposables à la fraude fiscale, à savoir la déchéance pour les entreprises concernées du bénéfice des différentes aides publiques, de quelque origine et nature fussent-elles, perçues par l'entreprise pendant les cinq dernières années accomplies. Il nous est en effet apparu que le maintien du bénéfice d'aides publiques pour des entreprises ne respectant pas les règles minimales de contribution aux charges communes ne pouvait se concevoir. On ne peut tricher d'un côté et continuer, de l'autre, de percevoir les subsides publics dont il est d'ailleurs à craindre qu'ils auront été, pour l'essentiel, détournés de leur objet. Au bénéfice de ces observations, je ne peux que vous inviter, mes chers collègues,

encore les difficultés financières de fraudeurs qui, à part quelques exceptions de personnes qui participeraient profondément à un système d'enrichissement personnel par ce système, essaient de tirer quelque profit d'un système de solidarité nationale.

de lutte contre la fraude mène un travail important, et je vous recommande, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, de l'auditionner. Sur le principe, madame la sénatrice, il y a un problème avec tous ces rapports.

que celle du texte adopté en commission. Par ailleurs, le texte adopté ne recouvre pas complètement la définition de l'article L. 111-7 du code de la consommation, puisqu'il ne prend en compte que l'un des deux alinéas. L'argument fondé sur le choix de fixer une définition d'opérateur de plateforme nous paraît faible. Notre groupe propose donc un choix pragmatique, qui évite tout risque juridictionnel. Quel

Monsieur le ministre, dans ce projet de loi, il manque bien évidemment l'essentiel. En effet, la disposition la plus efficace contre la fraude fiscale, c'est la baisse de la fiscalité dans l'un des pays les plus imposés au monde.

J'étais l'auteur du premier amendement que la commission a bien voulu introduire dans le texte. Il prévoyait une double transmission.

aux personnes qui vendent des biens d'occasion par internet leur numéro fiscal ? Surtout, quel est l'intérêt de transmettre ces informations à l'administration fiscale ? Selon moi, on engorge ainsi l'administration fiscale de données qui n'ont pas lieu d'être, puisqu'il n'y a pas d'imposition. Il vaudrait mieux demander aux

également de dissocier la vente par des plateformes des ventes au déballage. Il faut que les choses soient plus claires dans le code de commerce à cet égard. Pour ce qui concerne la fiscalisation, l'amendement renvoie à l'article 150 UA du code général des impôts. est l'avis de la commission ?

rapporteur, j'ajoute qu'il serait pour nous préjudiciable en termes de cohérence juridique d'introduire des exceptions non exhaustives au sein de l'article L. 110-1 du code de commerce qui définit l'acte de commerce. Par ailleurs, l'exception introduite portant sur les ventes par un particulier de biens meubles personnels et usagers nous semble trop large, puisque les ventes au déballage sont considérées en l'état du droit

une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales, après application d'un abattement de 3 000 euros. La mesure proposée crée des différences de traitement non justifiées par des différences objectives de situation et encourt, à ce titre, un risque de censure par le Conseil constitutionnel. En effet, la seule circonstance que des revenus soient perçus au travers d'une plateforme, et non pas directement, ne saurait justifier une différence dans le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu. La mesure conditionne l'avantage fiscal, c'est-à-dire l'exonération à concurrence de 3 000 euros, à une déclaration par la plateforme. Or le recours à un tiers déclarant ne peut pas justifier à lui seul l'exonération du revenu déclaré. En outre, le mécanisme créé par cet article ne concerne pas uniquement les petits revenus occasionnels et accessoires réalisés par des particuliers. En effet, l'abattement de 3 000 euros permet une exonération en faveur de toutes les entreprises, pourvu qu'elles exercent leur activité une plateforme. Toutes ces raisons ont conduit le Gouvernement à demander la suppression de cet article.

Selon les modalités de déclaration et selon le fait qu'on est adhérent ou non à un centre de gestion agréé, il y a 25 % de différence. Il faudra m'expliquer comment cela tient constitutionnellement. Sans doute est-ce lié à l'objectif de valeur constitutionnelle

Nous sommes réservés sur les articles qui viennent d'être adoptés, car les travaux en cours à l'échelon européen, notamment l'adoption du paquet e-commerce, nous paraissent de nature à répondre à beaucoup des préoccupations exprimées par le rapporteur, et ce dès 2021. La lutte contre la fraude à la TVA en matière de ventes effectuées au profit de particuliers à travers la plateforme d'e-commerce vient de faire l'objet d'une directive, le 5 décembre dernier. Ce dispositif harmonisé nous paraît constituer la réponse pertinente pour s'attaquer au problème de la fraude à la TVA dans le domaine soit des importations de biens à destination de consommateurs finaux, soit des ventes à distance intracommunautaires. Les nouvelles règles garantissent le paiement de la TVA dans l'État membre du consommateur final. Cela permet de consolider la nouvelle approche en matière de perception de la TVA dans l'Union européenne déjà en place pour les prestations de services électroniques et de respecter un engagement central de la stratégie pour un marché unique numérique en Europe. Par ailleurs, la directive prévoit que les plateformes de marché en ligne devront assumer la responsabilité de la perception de la TVA sur les ventes. J'ajoute que nous demandons aux plateformes de rendre publique et de communiquer sur l'identité des utilisateurs dès 2019 et d'assumer la responsabilité de perception sur les ventes réalisées sur leur plateforme par des sociétés établies dans des pays tiers auprès des consommateurs de l'Union européenne. Cela inclut notamment les ventes de biens déjà stockés par des entreprises de pays tiers dans des entrepôts au sein de l'Union, qui peuvent souvent être utilisés pour vendre frauduleusement des biens en franchise de TVA. Les nouvelles règles s'imposeront donc aux États membres, et la directive sera impérativement transposée pour une entrée en vigueur le 1 janvier 2021. La Commission a proposé une révision du règlement relatif à la coopération administrative en matière de TVA, qui contient aussi un certain nombre d'avancées positives de nature à faciliter les échanges entre les États membres, et ce avec le soutien unanime du conseil lors de l'Ecofin du 22 juin 2018. Dans ces conditions, l'instauration de dispositifs purement nationaux dans le domaine de perception de la TVA sur les opérations d'e-commerce ne nous semble pas souhaitable, ne serait-ce que parce que de tels dispositifs ne seraient pas en conformité avec la directive. Il nous paraît plus efficace de jouer collectif avec l'Union européenne. En outre, le dispositif mis à la discussion nous paraît moins opportun et moins robuste que la solution retenue par la directive e-commerce. Celle-ci rend redevable de la taxe la plateforme qui facilite les ventes au sein de l'Union, ventes réalisées par des non établis en Europe ou, plus largement, de toute livraison de biens importés d'une valeur intrinsèque de moins de 150 euros. Contrairement à la directive, le dispositif ne s'applique qu'à certaines plateformes, en l'occurrence celles qui ont plus de 5 millions de visiteurs par mois. Cela nous semble en réduire la portée. Par ailleurs, vous proposez un dispositif qui repose sur l'existence de présomption du non-respect des obligations par un redevable de la TVA, qui peut être établi non seulement en France, mais aussi n'importe où dans le monde. Nous pensons que cette exigence peut rendre le dispositif potentiellement peu efficace, voire inefficace lorsque la plateforme et le vendeur sont hors Union européenne. Et nous craignons également qu'il ne soit peu lisible, la notion de présomption n'étant pas définie. Sur le plan de la gestion fiscale, la mise en oeuvre d'une telle procédure nous paraît extrêmement complexe au 1 janvier 2019, qu'il s'agisse de la détection des plateformes concernées par le dispositif

Deuxièmement, il semble dangereux d'ajouter du travail à la commission des infractions fiscales, la CIF. Nous souhaitons quelle connaisse de davantage de dossiers à transmettre au pénal. C'est bien le sens de l'article 13.

Le problème est que cet article, à l'instar de son jumeau l'article 5, met une fois encore l'effectivité de la publication dissuasive en question, des voies de recours pouvant être sollicitées- cela se défend et se conçoit -, tandis que la commission des infractions fiscales se retrouve investie d'une nouvelle fonction : donner le feu vert à la publication des décisions de l'administration. Nous avons déjà souligné des problèmes très sérieux que posait l'existence de la commission des infractions fiscales du point de vue de la chaîne du droit dans notre pays. Cette commission sert de sas particulièrement sélectif au déferrement d'un certain nombre de contribuables au pénal.

des transactions éventuelles et des extinctions d'office ou presque de l'action publique ! Nous sommes donc partisans de ne pas saisir la CIF en cas de publication de décisions administratives. Au demeurant, celles-ci ont peut-être aussi le défaut de permettre une défausse sur toute procédure juridique potentielle.

sur la commission chargée d'autoriser ou non la publication des sanctions fiscales, instance qui est d'ailleurs une nouveauté. Le Conseil d'État a souligné qu'il s'agissait d'une protection

La commission des finances a adopté un amendement visant à ne publier que les sanctions devenues définitives. Nous pensons que le texte initial présente des garanties suffisantes. D'abord, toute décision de publication est prise après avis conforme et motivé de la commission créée.

de rendre publiables les sanctions uniquement après l'expiration de tous les délais de recours. Cela peut porter le délai de publication à plus de deux ans et faire perdre du sens à la sanction que représente la publication de celle-ci : rendre public le comportement délictueux. Par ailleurs, imaginons

part] à la préparation des dossiers à soumettre à la commission de publication des sanctions et à l'organisation des séances de la commission chargée de donner un avis sur les propositions de l'administration ; [d'autre part ] à la gestion des contentieux ». En revanche, pour les impacts budgétaires, il est écrit : « La publicité des sanctions prononcées par l'administration fiscale est de nature à prévenir la fraude fiscale et donc à augmenter les recettes publiques spontanément acquittées ».

recours du contribuable lui-même et celui de son conseil. Dans la rédaction actuelle, on pourrait tout à fait sanctionner un tiers, alors même que le contribuable,

le Gouvernement vise à renforcer les pouvoirs de l'administration fiscale dans la lutte contre la fraude fiscale, en sanctionnant les personnes proposant les montages frauduleux ou abusifs les plus graves, et non de simples schémas d'optimisation fiscale qui, eux, peuvent être parfaitement légaux.

préserve la liberté d'imagination des conseils, sans nécessairement en faire les complices actifs de ceux qui deviendraient ensuite, pour d'autres raisons et d'autres motivations, des criminels. En un mot, je défends le conseil

secrétaire d'État. Le Gouvernement considère que, en suspendant la possibilité pour les services fiscaux de sanctionner les tiers complices tant que la sanction appliquée aux contribuables n'est pas devenue définitive, le texte de la commission vide de sa substance la mesure proposée. Comme vous le

Ce délai de quatre ans pourrait, en effet, être largement écoulé à l'issue de la procédure contentieuse, rendant de fait impossible la sanction du tiers complice. On pourrait d'ailleurs On pourrait d'ailleurs sans peine envisager que des tiers complices conseillent à leurs clients d'engager des recours dilatoires, à seule fin d'échapper eux-mêmes à la sanction prévue à l'article 7. Ce n'est évidemment pas ce que nous souhaitons, les uns et les autres. Enfin, cet amendement,

dans le respect des principes généraux du droit, qu'il y a bien eu fraude fiscale. Sans cela, nous allons nous retrouver dans des situations ubuesques, violant tous nos principes généraux

ayant conduit à sanctionner un contribuable. La commission des finances a adopté un amendement tendant à restreindre les comportements à une liste définitive de prestations. Nous souhaitons revenir sur le caractère définitif de cette liste, avec un argument simple : réduire le champ de l'article conduira nécessairement à sanctionner moins. Nous sommes en l'espèce face à des avocats. Nous pouvons prendre le pari, aujourd'hui, que si nous restreignons cette liste, beaucoup prouveront avoir réalisé un autre type de prestations.

ils incluent, dans leurs coûts, les risques liés à ces sanctions. Nous pensons que, en termes d'efficacité et de dissuasion, il serait profitable de rendre ces intermédiaires solidairement redevables des pénalités fiscales. Cette disposition est

l'idée que l'intermédiaire intègre, comme vous l'avez imaginé, les coûts de l'amende à hauteur de 50 % du bénéfice dans son équilibre économique ne nous paraît pas un argument suffisant, pour une raison simple

demeure notifiant la pénalité soit contresignée par le directeur de l'organisme ou de la caisse lui-même, et non pas seulement par l'agent qui fait le contrôle et qui sanctionne. Ce contreseing est spécifié dans le code général des impôts ou dans le code de la sécurité sociale

Mme Sophie Taillé-Polian. Aujourd'hui, seule la notion de complicité permet de poursuivre pénalement les intermédiaires impliqués dans une fraude fiscale avérée. Cette notion nous semble donc limitée. limitée. Un rapport sénatorial préconisait de créer un délit spécifique d'incitation à la fraude fiscale comportant notamment la répression du démarchage et de la publicité pour des dispositifs d'évasion fiscale.

À cet effet, il a souhaité prévoir une sanction administrative contre des tiers, afin de compléter le droit en vigueur, qui permet, à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales contre un contribuable, de poursuivre le tiers complice. Ces instigateurs qui encouragent ou permettent la fraude encourent donc déjà, de ce fait, des sanctions pénales identiques à celles qui sont prévues aux présents amendements, voire supérieures en cas de circonstances aggravantes. Ces amendements ne sont par conséquent pas utiles, car la législation pénale existante permet de poursuivre et de sanctionner ces personnes. En revanche, l'article 7 du projet de loi complète le dispositif d'une sanction administrative qui vise la mise à disposition par les professionnels

qui, d'une certaine manière, légitiment l'amendement que nous avons déposé, au-delà des défauts éventuels de ce denier- vous connaissez notre modestie, maximal de l'amende encourue, actuellement 500 000 euros pour le délit de fraude fiscale simple- 2,5 millions d'euros pour les personnes morales -et 3 millions d'euros pour le délit de fraude fiscale aggravée- 15 millions d'euros pour les personnes morales pourrait désormais être porté au double du montant des sommes fraudées. Ce maximum légal alternatif paraît proportionné et justifié et n'appelle pas forcément d'observation en lui-même. Mais la moyenne des enjeux financiers des dossiers soumis à la justice pénale par l'administration fiscale s'établissant autour de 300 000 euros et le verrou de Bercy bloquant toute possibilité pour la justice de se saisir elle-même d'autres procédures plus importantes, la hausse prévue par le projet de loi n'aura qu'un impact finalement très limité. Le Syndicat de la magistrature relève d'ailleurs que le taux maximal actuel n'est en vigueur que depuis moins de six mois et qu'il est déjà proposé une nouvelle augmentation qui peut finalement apparaître comme soit de l'amateurisme, soit une opération de communication instrumentalisant la loi pénale dans le seul but de multiplier les effets d'annonce pour surjouer une certaine fermeté, mais qui n'aura finalement pas la moindre application concrète. Nous vous proposons donc, ce qui nous semble plus efficace,

collègue, vous proposez que les personnes condamnées pour fraude fiscale puissent également être condamnées à une interdiction de gérer une entreprise. Votre amendement nous paraît satisfait dans la mesure où l'article 1750 du code général des impôts prévoit déjà qu'une personne condamnée pour fraude fiscale

Il m'a semblé entendre dire, notamment au cours d'un certain nombre d'audiences qui traitaient de fraude fiscale, que des personnes, bien qu'elles aient été interdites de gestion, géraient quand même

explication de vote sur l'article.